Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur est reporté au mercredi 25 juillet à la suite de l'examen du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Acte est donné de cette demande. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

La principale hantise du propriétaire immobilier demeure le loyer impayé. En effet, on note une augmentation exponentielle de ce phénomène ces dernières années. Dans certains cas, la procédure d'expulsion qui en découle peut n'aboutir que trois ans plus tard. Pendant ce temps, le propriétaire ne perçoit plus de loyer, mais doit continuer à régler ses mensualités de crédit, les charges du logement et les frais liés à la procédure. Ces logements représentent bien souvent un complément de revenu indispensable pour les propriétaires. C'est pourquoi il est urgent d'encourager la location de logements en améliorant les garanties de paiement des loyers. À ce titre, le présent amendement vise à instaurer un prélèvement à la source des loyers par un organisme bancaire. en oeuvre sur l'initiative du propriétaire et permettrait aux deux parties de sécuriser le paiement du loyer. En effet, le locataire serait immédiatement prélevé de son loyer après la perception de ses revenus. Ainsi, il ne s'exposerait plus au risque de ne pouvoir honorer son loyer.

et les débiteurs de mauvaise foi ne pourraient plus générer de frais de relance supportés par le bailleur. Mais un locataire dans l'incapacité de payer est-il forcément de mauvaise foi ?

quand on est dans cette spirale, que l'on commence à ne plus pouvoir payer une facture, puis deux factures, puis trois, et quand commencent à s'accumuler des frais de dossier,

Il en est résulté un texte de consensus, qui transcende les clivages partisans, adopté à unanimité par le Sénat, et très attendu dans nos territoires. Nous avons aussi beaucoup dialogué avec vous, monsieur le ministre, et nos services avec les vôtres. Nous avons constaté un accord sur de nombreux points qui, aujourd'hui, figurent dans le texte de la commission. C'est que l'enjeu est essentiel. Il s'agit d'un enjeu de société : il suffit de circuler dans nos villes et villages pour constater l'état de dégradation et de souffrance dans lequel se trouvent nombre d'entre eux. Il s'agit aussi d'un enjeu politique, car il sera au coeur, n'en doutons pas, des prochaines élections municipales. Nous avons à présent l'occasion non seulement d'envoyer un signal politique à nos compatriotes sur nos priorités, mais aussi d'adopter des mesures concrètes. La commission des affaires économiques a apporté de substantielles et nécessaires modifications au texte gouvernemental. Celles-ci correspondent aux fruits du dialogue que nous avions noué et conclu avec vous, monsieur le ministre.

le Sénat : « Vous connaissez mon attachement au Sénat. Je suis donc très heureux de voir que la Haute Assemblée est, une fois encore, force de proposition en matière d'aménagement du territoire ». ». Vous ajoutiez : « il y aura débat à l'occasion de l'examen du projet de loi ÉLAN, dans lequel, d'ailleurs, je souhaite que nous puissions intégrer un maximum de ses dispositions ». « Maximum », le mot est fort ! Fort, mais imprécis Pour nous, en tout cas, il y a un « minimum », constitué du coeur des propositions de la commission. Et ce minimum, c'est d'abord l'article 54 F, mais ce sont aussi les articles 54 C, 54 H et 54 I. À cet égard, les amendements du Gouvernement sont extrêmement inquiétants et, à vrai dire, assez incompréhensibles. Le moment est venu pour le Gouvernement de montrer concrètement son intérêt pour le travail du Sénat et d'intégrer à son texte le « maximum » de ces dispositions dont vous nous parliez, monsieur le ministre, afin d'en faire un texte d'espoir pour nos territoires. Le moment est venu de savoir si notre dialogue aura été un jeu de dupes ou pas je vous remercie

Il était donc absolument normal, de mon point de vue, que le passage en commission imprime sa marque aux dispositifs prévus par ce projet de loi. Ainsi, le Sénat a affiché sa volonté d'aborder cette question sous un prisme différent. Le plan gouvernemental « Action coeur de ville » s'appuie sur une logique que l'on peut qualifier de « recentralisatrice » dans laquelle l'État sélectionne seul les collectivités réunissant les conditions pour être soutenues, laissant un trop grand nombre d'entre elles dans le besoin. À l'inverse, le texte issu des travaux du Sénat donne à tous les territoires, aux collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, un certain nombre d'outils leur permettant de mettre en oeuvre des solutions concrètes pour la revitalisation de leurs centres-villes et centres-bourgs, le tout en leur « laissant la main », puisqu'elle leur permet de garder la maîtrise de leur urbanisme et de leurs projets. C'est en ce sens que la proposition de loi sénatoriale est, à mes yeux, une réponse plus conforme aux attentes des élus locaux et des populations, et mieux adaptée à l'ensemble de ces enjeux. Il s'agit en effet d'une problématique majeure qui a conduit une revue, il y a quelques années, à parler de la « France moche », celle des zones industrielles ou commerciales en entrée de ville, celle de centres-villes désertés, à l'habitat vacant ou insalubre. Cette situation est le résultat de décennies d'effacement de l'État, d'abandon des territoires, de fermetures de services publics. Les enjeux sont donc multiples. Il faut tout à la fois que les collectivités locales obtiennent des outils et que l'État revienne dans ces territoires.

Nous mesurons le bénéfice de ces mesures, tout en considérant que c'est bien la logique globale qu'il faut changer. Il faut rompre avec ces politiques de gigantisme, d'étalement urbain inconsidéré, de mise en concurrence des territoires, des hommes et des entreprises, qui conduisent à la désindustrialisation et aux friches et, en définitive, à l'abandon des territoires fragiles et enclavés. C'est aussi la raison pour laquelle les pouvoirs publics doivent reprendre la main sur la finance : il faut remettre au coeur des politiques publiques la réponse aux besoins humains.

témoignant d'une véritable problématique que nous rencontrons toutes et tous dans nos départements, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs caractéristiques, et quelle que soit la diversité des villages et des petites villes de notre pays. nous avons évidemment soutenu cette proposition de loi. Pour autant, je crois qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que la revitalisation et le dynamisme des centres-bourgs et des centres-villes

Il nous a donc paru important d'agir, et de le faire de la manière la plus efficace possible. Je ne verserai ni dans les procès d'intention

pour coordonner des actions et flécher un certain nombre de crédits permettant aux villes moyennes d'accélérer la réalisation de leurs projets, voire d'en réaliser de nouveaux. J'entends parler de « recentralisation ». Drôle de recentralisation,

d'exiger de ces grandes structures- je ne citerai pas de noms -une contribution juste au développement de nos territoires.

Un certain nombre d'autres instruments peuvent également être mobilisés pour leur donner un coup de main. En outre, une collaboration est en cours avec un certain nombre de collectivités territoriales.

et de ne pas laisser les sociétés de conseil préempter les contrats. En effet, la logique de rentabilité financière qui, seule, gouverne ces cabinets serait insuffisante

éventail d'opérateurs d'assurer la mise en oeuvre des actions décidées par les collectivités locales. Je n'y vois pas de contradiction avec le texte de l'amendement ! Monsieur

cet amendement est surtout d'engager des procédures permettant la location-accession, donc de l'accession sociale progressive, pour contribuer à la mixité sociale dans les centres anciens.

faisant l'objet d'une ORT, en ouvrant la possibilité de déroger aux règles de densité, d'aires de stationnement et de gabarit prévues par le document d'urbanisme existant.

que son périmètre est automatiquement un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et un périmètre de mise en oeuvre du droit de préemption urbain

En l'occurrence, nous nous contentons de créer un droit automatique au profit des collectivités, lequel leur permettra, si elles le souhaitent, et seulement dans ce cas, de mobiliser deux instruments utiles de maîtrise du foncier sur leur territoire : le droit de préemption urbain renforcé et le droit de préemption commercial. Sans maîtrise du foncier, mes chers collègues, il n'y a pas de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs ! J'ajoute que cet élément de simplification a été adopté à l'unanimité par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Notre amendement vise à associer à toute ORT un processus d'évaluation simple, mais nécessaire. Sans cela, comment s'assurer que l'argent public est dépensé dans les meilleures conditions ?

La revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui font l'objet d'une opération de revitalisation de territoire, ORT, nécessite un tissu urbain réorganisé répondant aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes en matière de logement et de commerce. Ce tissu peut notamment comporter plusieurs dents creuses, non contiguës, et des secteurs non continus dans lesquels une action de revitalisation doit intervenir. Afin de permettre la réalisation d'opérations de restructuration d'ensemble favorisant la mixité fonctionnelle et la mixité sociale de ces espaces, cet amendement vise à autoriser, dans le cadre des ORT, la délivrance de permis d'aménager « multisites », qui constitueraient une alternative aux zones d'aménagement concerté. Dans ce cadre,

et d'entretien des voies, espaces et équipements communs liés à une opération d'aménagement multisites, mais aussi les situations de blocage susceptibles d'en résulter. Cette mesure de simplification tend toujours à s'inscrire dans une démarche expérimentale, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation du présent

nous tentons de sauvegarder les activités artisanales et commerciales maintenues dans les zones de revitalisation en cas d'installation de moyennes et grandes surfaces. tels projets, lorsqu'ils s'implantent dans le périmètre de l'ORT, ont un impact positif en matière de revitalisation du périmètre visé par l'opération de revitalisation territoriale, mais peuvent également constituer un facteur de déstabilisation pour les entreprises artisanales de proximité en exerçant des activités concurrentes, notamment dans le secteur alimentaire. Dès lors, si les objectifs poursuivis visant à faciliter l'implantation de nouveaux commerces en centre-ville sont évidents, il convient néanmoins de veiller à ne pas provoquer la disparition des activités commerciales artisanales existantes qui se sont jusqu'alors maintenues dans ces territoires et ont permis d'assurer la fourniture de services de proximité essentiels à la population. Il importe de rechercher des complémentarités entre les activités artisanales existantes et les projets d'implantation de moyennes et grandes surfaces en se fondant notamment sur des considérations d'aménagement du territoire ou d'équilibre concurrentiel. La limitation des dérogations aux projets inférieurs au seuil de 2 500 mètres carrés ne permet pas de garantir cette recherche de complémentarité. Même si les commissions départementales d'aménagement commercial n'ont pas donné entière satisfaction dans le rôle de régulateur qui leur a été confié, elles imposent la réalisation d'études d'impact fondées sur des critères d'aménagement du territoire, de protection des consommateurs et de développement durable. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l'alinéa 32 et, en conséquence, de l'alinéa 33

ou la réinstallation de locomotives commerciales dans les centres-villes. Depuis des années, ces locomotives ont plutôt eu tendance à s'installer en périphérie.

Les centres-villes ont besoin de locomotives pour restaurer leur attractivité. Cette disposition permettra d'assurer davantage de flexibilité aux élus pour aménager leurs centres-villes et adapter le dispositif d'exonération aux réalités de leur territoire. Là encore, cela s'appelle faire confiance aux collectivités territoriales.

à la condition que la commune concernée soit couverte par un document d'aménagement artisanal et commercial dans le cadre d'un SCOT ou d'un PLUI. L'objectif est de faciliter l'implantation de nouveaux commerces en centre-ville,

pour les entreprises artisanales et commerciales de proximité. C'est pourquoi le présent amendement vise à maintenir, pour les commerces alimentaires de plus de 1 000 mètres carrés, le passage en CDAC.

dans un centre-ville fragilisé. Il ne faudrait pas qu'une grande surface alimentaire, qui plus est d'une taille qui lui permette de regrouper des produits similaires, vienne détruire le tissu commercial existant.

est couvert par un DAAC qui organise les conditions d'implantation commerciale. En outre, je rappelle que le dispositif permet à la commune ou à l'EPCI de revenir à l'application

La revitalisation commerciale en centre-ville ne passe pas nécessairement par l'implantation d'une grande surface de vente à prédominance alimentaire qui peut, au contraire, entraîner un appauvrissement de l'offre de commerces de bouche ou des commerces artisanaux. Dans ces conditions, l'application d'un seuil plus bas, comme il est proposé dans l'amendement d'Élisabeth Lamure, pour ce type de commerce n'est pas illégitime. L'article L. 752-1 du code de commerce prévoit un dispositif particulier similaire en cas de changements d'activités des surfaces de ventes.

avons travaillé sur un type de CDAC qui reprendrait le modèle anglais. Elle effectuerait une étude préalable sur les impacts qu'aurait la création d'une grande surface non seulement sur la périphérie, mais aussi sur le centre-ville,

Je soutiens l'amendement d'Élisabeth Lamure, parce qu'il faut une limitation. Je ne me satisfais pas de voir revenir en centre-ville, sans limites et sans contrôle, les grandes surfaces qui ont vidé les centres-villes.

a souhaité revenir sur le caractère facultatif de la suspension par le préfet de l'examen des dossiers d'extension en CDAC, en intégrant les extensions d'ensembles commerciaux à la mesure de suspension.

est tenu de suspendre l'examen et l'enregistrement des autorisations commerciales des projets commerciaux s'implantant au sein d'une collectivité signataire de l'ORT, mais hors du secteur d'intervention. ailleurs, les suspensions d'autorisation ne se limitent pas au nouveau projet d'ensembles commerciaux, mais sont étendues aux extensions d'ensembles commerciaux. Conformément à l'avis du Conseil d'État, nous considérons que la suspension doit rester doit rester une faculté du préfet et non une mesure obligatoire, dès lors qu'il y a une demande de la collectivité. La décision du préfet doit être prise au regard du contexte local, en fonction des caractéristiques du projet, pour assurer le caractère limité et proportionnel de la mesure. C'est tout de même une avancée importante,

les extensions d'ensembles commerciaux à la mesure de suspension, alors que ces projets peuvent porter sur des modernisations, des mises aux normes d'équipements commerciaux vieillissants. Ces opérations seront soumises à autorisation dans les mêmes conditions

dans ces dossiers, renonçant parfois même à faire appliquer la loi. Il faut donc que les élus puissent obtenir des moratoires s'ils les jugent nécessaires.

l'enregistrement et l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale sans être saisi d'une demande. Par ailleurs, il permettrait qu'échappent automatiquement au moratoire, d'une part, les communes signataires d'une convention ORT, même si elles ne font rien concrètement, d'autre part, les communes d'un EPCI non signataire de la convention et non limitrophe. Les risques de contournement de la loi qui en résulteraient seraient considérables. Par ailleurs, dans bien des cas, des projets commerciaux de grande ampleur peuvent être davantage éloignés et avoir néanmoins un impact fort. L'amendement tend donc à permettre l'intervention du préfet sur sa propre initiative. d'ailleurs étrange de l'en empêcher ! Il vise à étendre au département le champ géographique potentiel d'un moratoire. Enfin, il a pour objet de clarifier et de simplifier la possibilité d'établir un moratoire dans le cas où un projet commercial risque d'avoir un impact excédant les limites d'un département. La responsabilité est confiée au préfet de région, au lieu de prévoir un arrêté conjoint de deux préfets de département, ce qui peut se révéler administrativement complexe, dans la mesure notamment où le pouvoir réglementaire sur une commission départementale ne peut relever que du préfet de département ou du préfet de région et pas du préfet d'un autre département, fût-il limitrophe. L'amendement n° 976 rectifié, présenté par M. Babary, Babary. Par cet amendement, il s'agit de répondre au besoin que peuvent avoir les opérateurs économiques d'anticiper les décisions de suspension des demandes d'autorisation d'exploitation, afin de ne pas construire inutilement des dossiers importants.

territoire. Il est donc proposé de compléter par l'avis de l'établissement public qui porte le SCOT les avis déjà donnés au préfet, quand celui-ci envisage de suspendre par

permettant au préfet de décider s'il doit ou non prononcer le moratoire. Or, depuis l'examen du texte par les députés, ces critères ont été clairement et objectivement définis. La commission estime donc que, dès lors qu'il apparaît, au regard de ces critères, qu'un projet est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de l'ORT, le préfet doit avoir compétence liée pour prononcer la mesure. Les termes « de nature à compromettre » sont très exigeants à cet égard pour l'analyse à laquelle il y aura lieu de se livrer. En outre, la mesure de suspension est tout aussi essentielle, qu'il s'agisse d'une création d'une surface de vente nouvelle ou d'une extension d'une surface de vente existante, car une extension importante est tout autant susceptible de compromettre la réalisation des objectifs d'une ORT qu'une création. S'agissant de l'amendement n° 255 rectifié la

et de ses effets sur la zone de chalandise. Or vous souhaitez que l'arrêté prononçant le moratoire soit préalable. Or il ne peut pas l'être. Quant à la notion de publicité « suffisante

au cas par cas », « projet par projet » du bien-fondé d'un moratoire, puisque le préfet devra analyser si un projet particulier « est de nature à compromettre les objectifs de l'opération ». Mais cela pourra conduire, le cas échéant, à ce que plusieurs projets puissent, eu égard à leurs caractéristiques propres, être soumis à un même moratoire. Les autres modifications proposées

pour des travaux effectués sur des logements existants qui n'emportent pas de création de surface de plancher supplémentaire. Il s'agit ainsi de répondre à la préoccupation très largement exprimée au travers d'un amendement de plusieurs de nos collègues, présenté en commission, et ainsi de favoriser la rénovation de l'habitat existant en zone tendue, notamment dans les centres-villes de villes moyennes, y compris dans ceux qui ne sont pas inclus dans le périmètre d'une ORT.

ne doivent se prononcer qu'à partir des pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En cas d'avis favorable, le porteur de projet produit les autres pièces nécessaires à la fin de l'instruction de sa demande de permis de construire. Cela permettra aux porteurs de projets de ne pas investir à fonds perdu d'importantes sommes d'argent dans les études et la conception des dossiers et aux administrations centrales de ne pas mener une instruction de permis de construire

et d'autorisation d'exploitation commerciale. Certes, cette procédure impose la réalisation d'un dossier complet de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, mais lorsque le projet est refusé uniquement au titre de cette autorisation, il ne peut pas

du permis, de ne pas retarder l'obtention du permis pour les projets ayant reçu un accord de la CDAC et, enfin, de limiter le nombre de demandes d'autorisation d'exploitation commerciale par des opérateurs sans motivation réelle à réaliser l'ensemble des projets

Quel est l'avis de la commission ?

l'on doit au ministre de la culture de l'époque, Jack Lang. Cependant, tous les gouvernements qui lui ont succédé n'ont jamais remis en question cette politique. C'est sans doute grâce à cela que l'on a encore en France des librairies indépendantes, qu'il faut, selon moi, soutenir. Par ailleurs, cet amendement ne coûte rien au budget de l'État. Il s'agit simplement de donner la possibilité aux collectivités qui le veulent d'accompagner ces librairies indépendantes. Pour ma part, je soutiendrai cet amendement, s'il est maintenu.

condamner les issues aux étages. Elles sont complétées par deux mesures réservées aux périmètres ORT, et la constatation automatique de l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble en cas de condamnation des accès.

de la situation des volets clos dans les centres-villes. Par ailleurs, cet amendement prévoit l'interdiction de travaux, qui obligerait, en pratique, de passer par le local commercial pour accéder aux étages. Cette interdiction est générale,

La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.

dès jeudi dernier, je vous ai interrogé sur l'affaire Benalla, devenue une affaire d'État. Les choses sont maintenant sérieuses. Nous ne saurions nous contenter de réponses dilatoires de votre part. Non, il ne s'agit pas de l'affaire d'un seul homme. Non, vous n'avez pas agi en temps et en heure.

Ce n'est pas acceptable ! Monsieur le Premier ministre, comme chef du Gouvernement de la France, allez-vous continuer à couvrir le silence du ministre de l'intérieur ? Notre peuple doit savoir : qui est M. Benalla ? Qui l'a recruté à l'Élysée ? Sur quel contrat ? Quel était son statut ? Quelles sont ses missions ? D'où vient-il ? Pourquoi de piètres sanctions, absolument pas proportionnées, malgré vos dires ? M. Benalla était chargé de la mise en place d'une officine de sécurité privée, ce qui pose la question de la confiance de l'Élysée à l'égard de notre police nationale. Pouvez-vous le confirmer ? Quels sont ses liens avec votre gouvernement, le ministère de l'intérieur ? les commissions d'enquête travaillent, mais vous avez le pouvoir de nous éclairer dès à présent. La crise est celle d'un régime hyperprésidentiel, d'un pouvoir jupitérien hors de contrôle.

et d'en finir avec la dérive monarchique qui est à la source de cette affaire. L'heure est grave, monsieur le Premier ministre. Vous devez au pays le respect et la transparence.

dans le fonctionnement de la commission qui s'apprête à procéder à l'audition de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur. Je ne doute pas que les membres de la commission des lois

je parle sous le contrôle de juristes, qui sont mieux formés que moi -n'est pas placée sous le contrôle de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et il y a des agissements, qui ne sont pas les agissements d'un individu,

Je ne suis pas là pour me prononcer sur ces copinages et sur les dérives auxquelles ils ont pu donner lieu. Mais je veux vous dire, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, que les actes

Je pense que cette mesure était proportionnée, mais je peux concevoir que vous contestiez cette affirmation, et qu'une discussion ait lieu sur ce point. C'est parfaitement légitime. Ce qui n'est pas, me semble-t-il, contestable, c'est qu'une décision et une sanction ont été prises rapidement. Et, de même, madame la présidente, dès lors que les faits ont été connus, l'ensemble des branches de notre démocratie, c'est-à-dire les trois pouvoirs, se sont saisies de cette affaire

Nous avons déjà tant appris ! Et quand l'ensemble des procédures seront suffisamment avancées pour que nous puissions en tirer des conséquences certaines et stables, alors moi, Premier ministre, chef du Gouvernement, je prendrai les décisions qui doivent

depuis la révélation de l'affaire Benalla, les plus hautes autorités de l'État sont confrontées à une crise politique majeure. Les faits égrenés et les premières auditions instruites par le Parlement montrent qu'il existe plusieurs graves dysfonctionnements au sommet de l'État. Je les énumère les sanctions disciplinaires prononcées ont été totalement inappropriées et, au demeurant, sans conséquence sur la place de M. Benalla dans l'organigramme de l'Élysée ; le ministre de l'intérieur et le préfet de police se contredisent dans leurs déclarations et rejettent sur les services de l'Élysée le fait de ne pas avoir dénoncé à la justice les faits délictueux dès qu'ils ont été portés à leur connaissance à leur connaissance ; le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, qui est aussi le premier responsable du parti majoritaire employeur d'un salarié directement impliqué dans cette affaire, le Président de la République reconnaît l'existence de dysfonctionnements, mais continue à s'enfermer dans un mutisme déterminé, accentuant le sentiment que les plus hautes autorités de l'État ont préféré protéger un individu qui leur est proche, quand il eût fallu protéger nos institutions. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, je ne veux pas me contenter de hurler au scandale ou de prendre la pose outrée : à chaque gouvernement son lot d'affaires et de polémiques. Mais, au regard des développements de ce dossier, je constate aujourd'hui que l'engagement réitéré du Président de la République de faire de la politique autrement est un faux-semblant où se manifestent des zones d'ombre et des arrangements. Je constate aussi que la gestion politique de cette affaire est le résultat de l'hypercentralisation du pouvoir exécutif, véritable contre-exemple de ce que nous devons faire en matière de réforme constitutionnelle. Monsieur le Premier ministre, comment entendez-vous renouer le lien de confiance avec les citoyens, afin de conforter notre République, qui est certainement « inaltérable », mais pas inébranlable ? Elle doit rester, en tout cas, irréprochable.

suis une fois de plus tombé dans un péché mignon. ce n'est pas une République qui serait composée d'individus, d'élus, d'hommes et de femmes, à tout jamais infaillibles. infaillibles. Ce n'est d'ailleurs pas ce que vous avez dit. Une République irréprochable, c'est une République qui regarde en face les dysfonctionnements, qui regarde en face ce qui ne va pas dans les comportements individuels,

caché les faits ! Les commissions d'enquête et la procédure judiciaire permettront- j'en suis certain -de décrire précisément l'enchaînement des faits

Nous vivons dans les institutions de la V République ; dans ces institutions, dans ce système parlementaire, le Premier ministre, le Gouvernement sont responsables devant le Parlement. C'est un fait, et c'est très bien ainsi. Le Président de la République, lui, n'est pas soumis à ce contrôle : ni lui politiquement, ni l'organisation de ses services. C'est un fait aussi, qui n'est pas neuf. Nous avons, ou plutôt nous avions, l'opportunité de discuter de ce sujet à l'occasion de la révision constitutionnelle. Et probablement, monsieur le président, vous et moi ne sommes-nous pas d'accord sur le sens qu'il faut donner à l'évolution de nos institutions.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir : M. Benalla voulait faire de la police sans que ça se sache, mais ça n'a pas marché J'espère que vous me pardonnerez cette entrée en matière ironique devant une situation très sérieuse, mais on ne peut manquer d'être frappé depuis quelques jours du contraste vertigineux entre, d'un côté, la farce d'une grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le « boeuf-carottes » et, le tourbillon politique qui met désormais en cause les plus hauts sommets de l'État et bloque les travaux de l'Assemblée nationale. L'une des raisons de cette situation, c'est un silence : celui du chef de l'État. Or ce silence devient pesant. En ne s'exprimant pas, non seulement le Président ne se protège pas, mais il s'expose. D'abord, il laisse les opposants les plus radicaux en situation de procureur, sans leur apporter de réponse définitive. Ensuite, il laisse se produire des contradictions entre les acteurs au cours de commissions d'enquête regardées par tous les Français, sans indiquer la voie du rassemblement. Enfin, l'anonymat des réseaux sociaux permet aux rumeurs les plus folles, les plus blessantes et les plus abjectes de proliférer sans aucun moyen d'y faire face. Le général de Gaulle disait que le Président de la République est en charge de l'essentiel. Il y a huit jours, l'affaire Benalla n'était pas l'essentiel ; aujourd'hui, que ce soit justifié ou non, elle l'est devenue. Il y a quinze jours, devant le Congrès, le Président proposait non seulement de pouvoir s'adresser aux parlementaires, mais aussi de pouvoir leur répondre. Aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement les parlementaires, mais de très nombreux Français qui attendent sa parole. Cette affaire, contrairement à ce que j'ai entendu, n'est évidemment pas le Watergate, ni même, pour rester en France, celle des écoutes de l'Élysée, le ou l'affaire des Irlandais de Vincennes. Mais en l'absence de réponse définitive, elle risque de devenir aussi délétère. Cette réponse claire et définitive, seul le Président de la République peut aujourd'hui l'apporter. Ce n'est donc pas une question que je vous pose, monsieur le Premier ministre, c'est une requête que je vous adresse : pouvez-vous lui dire que les Français attendent cette réponse ? La parole

de porter une appréciation sur une question qui est posée, il lui appartient d'y répondre. Permettez-moi de ne pas respecter ce principe et de vous dire combien les termes de la question que vous posez, l'humour dont vous faites preuve et l'élégance avec laquelle

le lieu et le message qu'il délivrera. Le 15 août ! Le moment venu, il exprimera ce qu'il considère devoir dire sur cette affaire. ! En attendant, le Gouvernement et moi-même nous répondons aux questions qui nous sont légitimement posées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous participons aux commissions d'enquête qui souhaitent auditionner les membres du Gouvernement et qui les interrogent avec rigueur et sans ménagement, ce qui est bien naturel. Nous faisons tout pour que le régime institutionnel de la V République, qui est parfois critiqué, critiqué, parfois porté aux nues, mais qui est le nôtre et qui est fondé sur cette particularité assez rare d'être un système parlementaire avec un président fort, fort, puisse continuer à fonctionner en reposant sur ses deux principes une présidence forte et un Gouvernement qui répond aux questions du Parlement et un Gouvernement qui répond aux questions du Parlement et qui est responsable devant lui. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour le groupe Les Républicains. Républicains. Monsieur le Premier ministre, il aura fallu moins d'une semaine pour que la France passe de la fête à ce climat opaque, pesant, dans lequel nous a plongés l'affaire Benalla. Cette affaire est-elle une affaire d'État ? Objectivement oui, car ce qui est en cause, ce n'est pas seulement un parcours individuel, celui d'un prétendu bagagiste, bagagiste, c'est beaucoup plus : c'est l'autorité de l'État ! Comment un proche du Président de la République peut-il se déguiser en policier pour passer à tabac des manifestants ? Au-delà, c'est le fonctionnement de l'État, de l'Élysée Comment cet individu, au passé déjà si lourd, s'est-il retrouvé au coeur du pouvoir ? Oui, il s'agit bien d'une affaire d'État, mais il s'agit aussi d'une affaire, monsieur le Premier ministre, qui concerne le chef de l'État. Tout ramène à lui : une ascension fulgurante, des privilèges exorbitants, une sanction trop indulgente ! Vraiment, oui, tout converge vers l'Élysée, et l'Élysée se tait, est mutique, contrairement à son habitude. Je reformule la question, que tous les Français se posent, monsieur le Premier ministre : quand le Président de la République sortira-t-il de son silence, quand prendra-t-il la parole pour s'expliquer devant les Français ?

Je constate que, à l'occasion de commissions d'enquête et de procédures judiciaires portant sur les faits qui ont eu lieu le 1 mai place de la contrescarpe, certains souhaitent évoquer des questions relatives à l'organisation de la présidence de la République, voire, le cas échéant, mettre en cause le rôle qu'aurait eu le Président de la République. Je ne suis pas sûr que cette évolution dans les questionnements repose sur une quelconque réalité.

le président, que la proportionnalité de la sanction prise par le directeur de cabinet du Président de la République était contestable. C'est une appréciation, qui est respectable et que je respecte, bien entendu, mais on peut ne pas la partager.

De même, dès que des faits nouveaux ont été rendus publics et connus- je parle de la transmission d'images que j'ai évoquée à l'occasion d'une question précédente

Pour le reste, je respecte les procédures qui sont engagées, notamment la commission d'enquête que votre assemblée a ouverte et les procédures judiciaires. Je ne peux pas me permettre de prendre des décisions de réorganisation ou visant à corriger des dysfonctionnements dès lors que je n'ai pas l'ensemble des éléments en ma possession. C'est d'ailleurs à ça que servent les procédures que vous avez vous-mêmes engagées. Aussi, monsieur le président, donnons-nous rendez-vous, au terme de cet exercice, pour que le Gouvernement- c'est sa responsabilité -puisse faire état devant le Parlement des décisions qu'il prendra à la suite de cette affaire. Monsieur le Premier ministre, si je vous comprends bien, finalement le Président de la République se serait vu imposer à ses côtés, dans son intimité, la présence de M. Benalla ! Cette affaire est révélatrice. Un pouvoir qui prétend récapituler, résumer, incarner ou réincarner l'essentiel de tout l'édifice républicain, au mépris des contre-pouvoirs, des corps intermédiaires, un pouvoir qui s'isole, un pouvoir solitaire devient inéluctablement un pouvoir arbitraire. Il se voit au-dessus de tout, il ne se sent tenu de rien. Eh bien, monsieur le Premier ministre, tirez les leçons de cette affaire modifiez le projet de texte constitutionnel. Nous n'avons pas besoin que la Constitution place encore plus de pouvoirs dans les mains d'un seul. La République est fragile, elle n'est pas inéluctable. À vous de la préserver !

le comportement d'un chargé de mission à la présidence de la République occupe l'ordre du jour parlementaire depuis plus d'une semaine. C'est fort, peu d'entre nous y arrivent

Laissons-les cheminer et attendons leurs conclusions. Je reviendrai à mon tour sur le rôle et l'effet institutionnel de cette affaire. C'est un peu l'effet papillon.

l'affaire dont nous parlons aujourd'hui était à l'ordre du jour du Parlement depuis plus d'une semaine : c'est inexact. Permettez-moi, du reste, de souligner

et l'enseignement qu'il faut tirer des circonstances. C'est une règle simple, que je m'assigne depuis que j'ai commencé à travailler, d'essayer de faire en sorte que tout ce qui arrive ou que tout ce qui m'arrive

il n'y aurait pas pire législateur, et probablement pas pire gouvernant, que celui qui renoncerait à apprendre, à prendre en compte les éléments nouveaux dans sa réflexion. réflexion. Tout cela doit-il nous conduire à renoncer à la révision constitutionnelle telle qu'elle a été proposée par le Président de la République et telle que le Gouvernement

Je ne le crois pas. Je pense que c'est un bon débat, je pense que c'est une bonne réforme, je pense qu'il est utile de la discuter au fond. Elle est, comme vous le savez, composée de trois textes : un projet de loi constitutionnelle, un projet de loi ordinaire, un projet de loi organique. Nous n'avons pas pu aller au terme de l'examen du projet de loi constitutionnelle. Il nous reste la possibilité, soit de recommencer à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi constitutionnelle, soit le cas échéant de passer aux deux autres textes. Cette possibilité est techniquement ouverte. Je n'ai pas tranché.

» ? Ayons un peu de nuance aujourd'hui et faisons le savoir. Après les outrances, les manipulations et les interprétations hasardeuses, prenons un peu de recul et de hauteur face à la réalité de ce qui est non pas une affaire d'État, mais une grave dérive individuelle et un comportement inacceptable. Beaucoup de responsables cherchent à opérer une récupération politique en se drapant dans la vertu et l'angélisme, attitude qui, vous le savez bien mes chers collègues, conduit au populisme. Ce sont des De façon unanime, nous affirmons clairement la gravité des faits qui sont avérés. Nul n'est au-dessus des règles et des lois : il n'y a pas eu, il n'y a pas et il n'y aura pas d'impunité.

Nous affirmons qu'il n'y a ni police parallèle ni milice privée. La commission d'enquête a reçu notre approbation. Nous voulons que les Français soient totalement informés et que cesse ce déchaînement de haine, d'anathèmes et d'imprécations. Monsieur le Premier ministre, le Sénat prend ces événements avec recul et modération. Notre chambre assume toute sa fonction et son rôle de législateur et de contrôle du Gouvernement, et fait preuve de responsabilité en poursuivant l'examen des textes. Là n'est pas la question ! Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer que l'épreuve que nous traversons actuellement n'empêchera pas le Gouvernement de poursuivre les réformes engagées, notamment celle que vous avez évoquée tout à l'heure

nul n'est au-dessus des lois. Ce principe simple, mais essentiel, est la garantie que nous vivons dans une démocratie. Nul n'est au-dessus des lois

de quoi que ce soit, même ceux-là ne sont pas au-dessus des lois, et c'est tant mieux ! Je suis déterminé, avec l'ensemble du Gouvernement- je l'ai dit tout à l'heure, je le redis bien volontiers tirer toutes les conséquences des enseignements que nous pourrons dégager des procédures qui ont été engagées afin d'éviter que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent. De la même façon, l'ensemble du Gouvernement est déterminé à mettre en oeuvre les engagements qui ont été pris par le Président de la République devant les Français. Si pendant quelques jours, à l'Assemblée nationale, le débat a été impossible, si pendant quelques jours on a voulu faire d'une dérive individuelle quelque chose qui relèverait d'une affaire d'État, ce que je conteste formellement, je tiens à dire ici avec fermeté et tranquillité, mais avec détermination, que rien ne nous fera dévier du projet présidentiel. Nous mettrons en oeuvre les engagements qui ont été pris par le Président de la République devant les Français pour réparer notre pays et pour faire en sorte d'en faire le pays le plus attractif, le plus compétitif et le plus sûr.

la presse a joué son rôle de lanceur d'alerte. Des faits graves ont été mis sur la place publique, des imputations personnelles avancées, des allégations répétées. L'Assemblée nationale exerce son contrôle. Le Sénat aussi, mais avec sa propre tonalité, en inscrivant son investigation dans un périmètre plus large. Nous faisons toute confiance à notre commission des lois pour faire la lumière sur les faits allégués et les responsabilités personnelles, dans la sérénité et le plus strict respect de la séparation des pouvoirs. Quant à la justice, elle se prononcera le moment venu. Pour autant, la situation que nous connaissons survient à un moment particulier, celui de la réforme de nos institutions voulue par le Président de la République. Une réforme dont l'examen a été reporté à l'Assemblée nationale. Dans ce qui ressemble à une mise en abîme, nous avons pourtant sous les yeux la démonstration que notre démocratie a besoin d'un équilibre raisonné des pouvoirs, avec un Parlement moderne et fort, qui exerce pleinement sa mission de législation et de contrôle. Dans ce schéma, le Sénat a bien sûr toute sa place en tant que contre-pouvoir constitué et responsable, comme il l'a toujours été. Ce qui importe surtout, c'est que les dérives d'un individu ne fassent pas le lit de la démagogie et des populismes, qui avancent à découvert et sans ambiguïté. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer la nature des évolutions à apporter à la révision constitutionnelle et les éléments qui fonderont votre décision ?

la confiance que vous exprimez dans les institutions de notre pays, le souci de faire en sorte qu'elles puissent jouer leur rôle le plus complètement possible et que nous puissions tous, quelles que soient nos responsabilités, en tirer les conséquences pour prendre de bonnes décisions et éviter que des dysfonctionnements ne se reproduisent. Je partage en tout point aussi l'idée selon laquelle il ne faut pas confondre les rôles et qu'il faut- c'est d'ailleurs une des garanties de la démocratie -faire en sorte que les procédures puissent aller librement à leur terme.

à la fois pour des raisons liées à l'équilibre des pouvoirs- on peut très bien l'entendre -, mais aussi parfois pour des raisons liées à une opposition de principe aux propositions contenues dans ce projet de révision constitutionnelle.

ce projet à la discussion parlementaire, en application des dispositions de l'article 89 de la Constitution. Nous ne changeons pas de logique. il nous faudra évidemment prendre en compte cet élément nouveau dans la définition du calendrier de travail de la rentrée, aussi bien à Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on peut faire de chic, car, vous le savez, la deuxième partie de l'année est incroyablement occupée par les questions liées notamment à l'examen et au vote du budget. Il faudra donc que nous trouvions le bon moment pour présenter le ou les textes qui s'inscrivent dans ce projet de révision constitutionnelle, et je suis heureux de savoir que, le moment venu, ce débat aura lieu. Jean-Claude Requier, pour la réplique. Le temps médiatique n'est pas le temps parlementaire. Le rythme sénatorial n'est pas rythme de l'Assemblée nationale. Ne cherchons donc pas à coller au flot de l'actualité, au sensationnel et au renouvellement incessant de l'information. Écartons l'émotion et l'agitation. Gardons plutôt la sérénité, la réflexion et la sagesse, qui sont la marque de notre Haute Assemblée.

de l'État. Elle a révélé l'existence d'un très proche collaborateur, puisqu'il s'agit du chef adjoint de cabinet du Président de la République, au comportement aussi étonnant qu'inacceptable dans notre État de droit. Par son attitude, cette personne a jeté inutilement l'opprobre sur nos services de police et sur le fonctionnement des dispositifs de sécurité du Président de la République. M. le ministre de l'intérieur a été interrogé et auditionné hier à l'Assemblée nationale. Il le sera dans quelques minutes au Sénat devant nous et nous attendons de sa part des précisions sur les déclarations qu'il a déjà fournies. M. le préfet de police a lui-même répondu hier à cette commission d'enquête avec clarté et précision, ce que nous soulignons. Nous apprenons de ces différentes déclarations que des mensonges ont été

La commission des lois fera son enquête pour révéler les failles de ce dispositif incroyable. Il n'empêche qu'une question subsiste : alors que ce très proche collaborateur le Président de la République, avec des compétences fortes et un pouvoir énorme au coeur de la République, est en cause, pourquoi le Président ne dit-il rien, pourquoi ne parle-t-il pas ? Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur François-Noël Buffet, nous nous connaissons depuis quelque temps et je pense que vous me savez homme d'honneur. Tout à l'heure, devant votre commission, je témoignerai en disant, selon le serment qui est prêté, la vérité, toute la vérité ! Oui, cette histoire est une histoire tragique,

est venu sur une opération sur laquelle il n'aurait jamais dû aller, en tout cas jamais dû aller tel qu'il est allé, non pas en tant qu'observateur, ce qui est possible pour chacun d'entre nous,

Le directeur de cabinet du ministère de l'intérieur s'est enquis auprès du directeur de cabinet du Président de la République pour savoir s'il condamnait ces faits.

quelques secondes. Le Président s'est enfermé dans le silence. Mais ce silence distille tous les jours un poison insupportable pour l'État et pour la République. La parole est à M. Alain Richard, pour le groupe La République En Marche. Quelques défis économiques et sociaux continuent d'interpeller notre pays.

Je comprends qu'ils ont établi un programme de travail visant à l'adoption de plusieurs accords collectifs traitant

de ces différentes opérations de concertation et de négociation, et comment, puisque je vois que M. le secrétaire d'État Christophe Castaner me répondra, dans le cours des travaux de réforme sociale, le travail avec les partenaires sociaux pourra également être communiqué et dialogué avec le Parlement Richard, il est essentiel de porter une attention et une confiance particulières au dialogue social. Cela a été une constante, sous l'autorité du Président de la République du Premier ministre Édouard Philippe, depuis un an. Et si la forme a évolué, avec le choix d'une réunion multilatérale, cette rencontre s'inscrit dans la continuité des échanges entre le Président de la République et les partenaires sociaux.

les rencontres avec les partenaires sociaux ont été constantes. Là encore, le dialogue existe, même si, à un moment donné, on peut constater des désaccords et si chacun, dans le cadre de ses responsabilités, doit décider. Lors de cette rencontre avec le Président de la République, la matinée a été consacrée à des échanges constructifs autour des réformes qui seront engagées dans les prochains mois sur le champ du travail. Avec les partenaires sociaux, il a été convenu de travailler : premièrement, sur la modernisation de l'action publique et la rénovation du paritarisme dans le cadre d'une République contractuelle deuxièmement, sur l'inclusion et la lutte contre les discriminations ; troisièmement, sur les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Cette volonté de travail s'étend aussi à l'agenda international. La France accueillera et présidera le G7.

Une phase de négociation est nécessaire, une phase de discussion s'ensuivra. Il est évident aussi que nous devons, au-delà de ce seul sujet, travailler sur l'articulation entre les prestations d'assurance et la solidarité dans le champ de l'indemnisation chômage. Plusieurs organisations ont fait part de leur volonté de se saisir de cette négociation après une phase de négociation partagée. Il faut conclure. Bien évidemment, le Gouvernement sera attentif à ce travail et à cette discussion partagée.

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre, mais je n'aurai pas droit à sa réponse. Monsieur le secrétaire d'État Benjamin Griveaux, vous répondrez à sa place. Tous les éléments qui ressortent des investigations menées par la presse dans l'affaire Benalla et toutes les auditions, mes chers collègues, qui ont eu lieu hier à l'Assemblée nationale ont un point commun c'est vers l'Élysée que les regards se tournent, vers son premier locataire. Il y a quelques mois, pendant la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron déclarait devant les Français lors d'une grande émission : « Dès qu'il y a une bavure, il doit y avoir une réponse et une sanction Mais elle est hiérarchique ... Je crois, moi, à une République de la responsabilité. » Propos plein de sagesse du candidat, que le Président semble avoir oublié ! Depuis plusieurs jours, le Président de la République, d'ordinaire si bavard, devient taiseux. Je me pose cette question. On voit se dessiner une stratégie, la stratégie silencieuse du Président de la République : échapper à sa responsabilité et trouver parmi ceux qui sont sous son autorité directe des boucs émissaires. En préparant ma question, je me souvenais de la définition qu'Antoine de Saint-Exupéry donna du chef : « Le chef est celui qui prend tout en charge. Il dit : " J'ai été battu ". Il ne dit pas : " Mes soldats ont été battus " Monsieur le Premier ministre, monsieur le secrétaire d'État Benjamin Griveaux, un chef doit assumer ! Pouvez-vous nous dire où est passé le Président de la République ?

Ici, on s'attache aux faits. Quels sont les faits, à ce jour, établis ? Car, certes, il y a la parole, mais il y a aussi l'action. L'Élysée a agi rapidement : dès le 3 mai dernier, des sanctions ont été prises à l'endroit de M. Benalla. Une procédure de licenciement a été engagée le 20 juillet à son endroit. Le Président de la République a confié au secrétaire général de l'Élysée l'analyse des dysfonctionnements, afin de pouvoir y remédier et de faire des propositions de réorganisation, pour que des dérives comportementales individuelles ne puissent plus se produire à l'avenir. Depuis quatre enquêtes ont été ouvertes : une enquête administrative, une enquête judiciaire et deux enquêtes parlementaires, dont l'une va s'ouvrir prochainement dans cet hémicycle. Vous m'interrogez sur la parole du Président de la République. Loin de moi l'idée de parler au nom du Président ou à sa place. Mais permettez-moi de partager une observation avec vous, madame la sénatrice. Il me semble que, depuis une semaine, le Président de la République a préféré être le garant impartial de nos institutions, plutôt que de céder aux artifices de la communication. Qu'aurions-nous pensé, collectivement, d'un Président de la République qui serait intervenu dans le débat public ? Nous aurions dit- et nous aurions eu raison de le faire ! -qu'il interférait et qu'en cela il n'était pas le garant de nos institutions et de la séparation des pouvoirs auxquelles, je le sais, vous êtes attachée, madame la sénatrice, comme y sont attachés l'ensemble des sénateurs sur ces travées.

et c'est sa marque de fabrique, on ne cherche pas à faire payer ses collaborateurs. On affronte ses erreurs et on prend ses responsabilités ! La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour le groupe socialiste et républicain. Ma question socialiste et républicain. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale. Je ne vais pas parler de l'affaire Benalla, mais des 22 millions de nos concitoyens, dont 3 millions d'enfants, qui ne partent pas en vacances, soit 36 % de la population. Cette situation est celle de la France en 2018, et c'est inacceptable. Ainsi, un tiers des 15-24 ans, une personne handicapée sur trois ou encore un enfant issu d'une famille d'ouvriers sur deux n'ont pas accès aux vacances. Précarisation croissante des ménages les plus modestes, chômage des jeunes, baisse des aides on assiste depuis plusieurs années à un recul de la réalisation du droit aux vacances, un droit pourtant inscrit dans plusieurs textes, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce droit est fondamental, notamment pour la jeunesse. Il est facteur d'inclusion sociale et d'épanouissement, mais c'est aussi un enjeu de santé publique et un apport économique indispensable. Les vacances font partie du cursus éducatif. C'est déjà l'apprentissage de l'autonomie et du vivre ensemble. Je souhaite saluer l'engagement des associations d'éducation populaire, et notamment du Secours populaire, qui font un travail remarquable et permettent à de nombreux enfants issus de familles modestes de partir en vacances une fois dans l'année. Dans la Drôme, par exemple, la Fédération des oeuvres laïques permet à 1 200 enfants de partir en colonie de vacances. Mais cette année, avec la diminution drastique des contrats aidés et la mise en place trop tardive des parcours emploi

? Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il mettre en place pour lutter contre ces exclusions et intégrer davantage le droit aux vacances dans les politiques familiales, sociales et de jeunesse ?

concernant le départ des enfants en vacances. Ce problème n'est pas nouveau. Vous l'avez rappelé, si l'on regarde l'évolution depuis le début de la décennie, il y a beaucoup moins d'enfants qui partent en colonie de vacances chaque année. Il faut donc s'interroger sur ce phénomène au plan tant quantitatif que qualitatif. Environ 1,5 million d'enfants partent en colonie chaque année. Ils étaient 300 000 de plus au début de la décennie.

que nous regroupions davantage les moyens publics et privés, ceux des collectivités locales et de l'État, afin de pouvoir mener une action sociale vis-à-vis des enfants. Cela commencera l'année prochaine, avec le plan Mercredi, qui traduit un nouvel élan du périscolaire. Nous mettrons plus de moyens, avec les caisses d'allocations familiales en particulier, pour les activités périscolaires des enfants le mercredi. Cela continuera avec les activités extrascolaires et les vacances. Je m'y engage.

Pour rappel, la législation applicable aux préenseignes installées le long des routes et aux abords des communes a été récemment réformée, en 2010, afin de préserver la qualité des paysages, le cadre de vie et l'environnement. D'ailleurs, la commission de la culture de notre assemblée a été particulièrement en pointe sur ce dossier. Ainsi, ce dispositif a été interdit aux activités susceptibles d'intéresser les personnes en déplacement, l'hôtellerie et la restauration en particulier. Or les députés ont introduit par voie d'amendement une dérogation pour les restaurants, qui pourraient par conséquent de nouveau installer des préenseignes, aux entrées de ville notamment. Ce retour en arrière n'est pas souhaitable pour plusieurs raisons. Premièrement, la multiplication de ces préenseignes, disposées souvent de manière anarchique, crée une forme de pollution visuelle qui nuit à l'attractivité des territoires, que ce soit en milieu urbain ou rural. Nous avons tous en tête l'image de ces panneaux, parfois plantés en plein milieu des champs ou dans d'autres espaces improbables. Deuxièmement, de nombreux efforts, y compris financiers, ont été effectués par les élus locaux afin de substituer à ces préenseignes d'autres dispositifs d'information des usagers, beaucoup plus respectables du patrimoine naturel, voire du cadre de vie urbain. Rétablir une dérogation au droit actuel serait finalement faire fi de cet engagement, ainsi que du travail réalisé. Enfin, une telle disposition peut s'avérer contraire à un objectif unanimement poursuivi sur les travées de cette assemblée, en l'occurrence- nous en avons parlé précédemment -, la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes, concrétisée dernièrement par l'adoption de la proposition de loi de nos collègues Martial Bourquin et Rémy Pointereau. En effet, étant précisé que beaucoup de ces préenseignes de restauration concernent des établissements situés à la périphérie des centres-villes ou des bourgs, favoriser une dérogation en la matière reviendrait à porter un préjudice à leur attractivité. Ainsi, après avoir oeuvré à leur redynamisation, il serait particulièrement dommage de voter un article allant à l'encontre de cette finalité. Mes chers collègues, si les enseignes et autres panneaux peuvent, on le sait, avoir parfois de véritables vertus, je pense qu'en l'espèce il conviendrait d'être prudents et plutôt raisonnables en en maintenant en l'état le droit actuel.

Les communes et les départements ont mis en place d'ambitieux plans de signalisation d'information locale, la SIL, pour interdire les préenseignes sur les routes et les abords des communes, afin de préserver l'esthétique de nos paysages et nos communes ruraux. L'article 54 A est un retour en arrière par rapport à ce travail, mené et accepté majoritairement par nos collectivités, pour éviter la publicité anarchique.

pour présenter l'amendement n° 652 rectifié. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a été à l'origine de la réforme de la législation applicable aux préenseignes, opérée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, qui a conduit à restreindre le champ des activités susceptibles de faire l'objet de préenseignes, et en particulier à interdire ce dispositif pour signaler, entre autres, les lieux de restauration. Plusieurs arguments ont été à l'origine de cette évolution : les fortes nuisances causées par la multiplication et l'installation anarchique des préenseignes le long des axes routiers, au niveau des entrées de ville et au milieu des champs, et leur impact sur les paysages, particulièrement sensible en milieu rural le difficile contrôle des préenseignes par les maires, en raison de leur positionnement fréquent à la lisière des territoires des différentes communes. Une proposition avait été faite et offerte en 2008 mettre en place des équipements d'enseigne à proximité de la voirie, sans dénaturer les paysages, regroupant sur un même panneau de dimensions réduites les différentes mentions concernées. Ces arguments, qui n'ont pas évolué depuis 2010, plaident en faveur de la suppression de l'article 54 A, qui prévoit une dérogation pour la restauration. Lors du débat à l'Assemblée nationale, vous avez dit, monsieur Denormandie : « Il ne faudrait pas, en essayant de résoudre le problème, ouvrir la vanne

liées à cet article, a dit préférer que cette décision soit adoptée, même non juridiquement « calée », et faire confiance à la sagesse des sénateurs pour corriger et affiner la rédaction. Il y a là un sujet pour la restauration en secteur rural, nous en convenons tous. Mais cette mesure a de nombreux effets pervers, notamment pour la qualité de nos paysages. Elle favorise aussi une concurrence qui est nuisible à ces fameux restaurants que nous voulons défendre et aider. Monsieur le ministre Mézard, lors de ce même débat, vous avez dit : « Il n'est pas non plus dans l'intérêt des propriétaires de ces restaurants de saccager le patrimoine et les paysages ruraux. » Il me semble que, faute de s'être donné le temps d'évaluer cette mesure, de conclure à une taille de commune pour laquelle la dérogation pourrait être acceptée, de traiter de chartes paysagères et de leur contenu, faute d'avoir travaillé ces questions dans de nombreux EPCI autour d'un règlement local de publicité et de normes éventuelles, bref, faute d'avoir pris le temps d'un travail sérieux, la sagesse serait

dont le dispositif n'opérait qu'une extension très limitée du champ des préenseignes aux activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir,

à deux objectifs qui peuvent paraître, au moins en partie, contradictoires : d'un côté, la nécessaire préservation

avait donné lieu au Sénat à de longs débats contradictoires et provoqué une levée de boucliers dans les territoires de la part, évidemment, des restaurateurs, mais aussi des élus locaux. L'évolution de la réglementation à laquelle est fait allusion n'est qu'un palliatif qui a été mis en place pour essayer de contrebalancer cette décision. Bien sûr, je sais que d'autres professions, comme les artisans et les garagistes, demandaient

pour explication de vote. Si je peux comprendre certaines prises de position, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aussi savoir tirer les leçons de certaines erreurs.

Ces pertes sont significatives puisqu'elles peuvent aller jusqu'à une baisse de 25 % du chiffre d'affaires. Le retrait des préenseignes pénalise donc nos zones rurales déjà fragilisées et, surtout, les petits établissements qui n'ont pas ou plus de moyens d'information et de signalisation pour la clientèle de passage. L'article 54 A a rétabli les enseignes indispensables à ces restaurants ruraux- je parle bien des restaurants ruraux -, sans pour autant risquer d'en faire bénéficier

M. le ministre a expliqué que le débat avait été long et charpenté à l'Assemblée nationale ; je veux rappeler que le débat avait été aussi long, charpenté et très argumenté au

ont constaté que, même s'ils sont présents sur les réseaux sociaux, ils ont perdu beaucoup de clientèle. L'Assemblée nationale, à mon avis, a fait preuve de sagesse en introduisant l'autorisation d'installer des préenseignes pour les restaurants.

le fruit du travail de ceux qui y vivent. Le jour où plus personne n'y vivra, on pourra s'extasier devant des paysages qui seront totalement vides

les dérogations pour l'installation de préenseignes, mais pas seulement pour les restaurants. Il s'agit non pas du tout de défigurer les paysages, mais plutôt de donner une bouffée d'oxygène à des territoires ruraux qui sont en souffrance parce qu'ils manquent de visibilité.

Informer de la présence non seulement d'un restaurant, mais aussi d'un café, d'une auberge, d'un hôtel, d'activités artisanales ou commerciales me semble être le seul moyen, dans certains cas, pour permettre à des villages, à des zones de continuer à avoir une activité. L'aménagement du territoire, c'est aussi l'activité économique. Même si la présidente

hors agglomération, en restreignant certaines activités susceptibles d'en bénéficier. Pour certaines activités, les préenseignes ont été remplacées par la signalisation d'informations locales- cela a déjà été évoqué -, mais cette dernière s'avère peu lisible, notamment pour les automobilistes hors agglomération, et donc inadaptée aux activités liées au tourisme, en particulier en milieu rural. Ainsi, les activités de restauration et d'hébergement ont été particulièrement touchées par cette nouvelle réglementation, avec une perte moyenne de 25 % de leur chiffre d'affaires. Pourtant, la survie de certains établissements qui assurent un rôle social et économique incontournable et majeur dans nos territoires ruraux dépend effectivement d'une préenseigne les signalant à la bifurcation, notamment, d'un axe ou d'axes principaux de circulation. Malgré l'essor du numérique, un grand nombre d'automobilistes, en particulier la clientèle de passage, a besoin de voir un panneau indiquant un hôtel, un restaurant ou un bar. Adopté par l'Assemblée nationale, l'article 54 A prévoit d'élargir la dérogation aux restaurants vendant des plats fabriqués à partir de produits du terroir. Sans remettre en cause la préservation de nos paysages ruraux, il est proposé d'élargir les préenseignes dérogatoires hors agglomération à l'ensemble des activités de restauration et d'hébergement, en soutien à l'économie rurale. L'amendement n° 1035 rectifié,

Des exceptions ont été admises, sous conditions, à l'intérieur de l'emprise des aéroports ou des gares, ainsi qu'à proximité des centres commerciaux. Les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales font l'objet d'une tolérance. Les députés ont souhaité étendre cette dérogation à l'ensemble des restaurants qui proposent de tels produits. Par le présent amendement, il est proposé d'introduire une nouvelle entorse au principe évoqué, en ciblant particulièrement l'hôtellerie de plein air. En effet, les préenseignes sont essentielles pour les campings, à la fois pour mieux les localiser

aussi intéressant que celui-là ? Pourtant, la durée de vie d'une telle enseigne dans une commune de 2 500 habitants peut être relativement limitée. L'opticienne avait installé trois panneaux à l'entrée du village qui permettaient de mettre en avant son activité.

Lorsqu'il y a des préenseignes ou des enseignes sur un territoire, cela veut dire que le territoire va bien. Le jour où il n'y en aura plus, ce sera très grave.

montré l'évolution de leur activité économique. On a expliqué, tout au long de nos débats, qu'il fallait faire preuve d'écoute, de respect et de pragmatisme.

de déduction fiscale qui incite les propriétaires à mettre en location leur logement à un loyer de montant intermédiaire, social ou très social. Plus le loyer pratiqué est abordable et le logement situé dans une zone où il est difficile de se loger, plus la déduction fiscale est élevée. Actuellement, ce dispositif est mobilisable en zone C uniquement pour de l'intermédiation locative. Les évolutions proposées pourraient être de nature à renforcer l'attrait de ce dispositif, qui, en lui-même, n'a que des côtés positifs, et à en faire un outil d'accompagnement à la revitalisation des centres-villes.

soit 8,4 % du parc immobilier. Dans certaines villes, ce taux s'établit même à 10 %. Il est donc prioritaire d'agir sur cette vacance. Le dispositif de l'intermédiation locative est l'une des réponses à cette difficulté. Il permet de capter des logements privés et de les prendre à bail pour loger des personnes aux revenus modestes. Le principe en est simple : une association est locataire d'un logement privé, qu'elle sous-loue à une personne contre un loyer compatible avec les moyens de celle-ci, tout en assurant l'accompagnement social.

Pour inciter les propriétaires à confier leurs biens à l'intermédiation locative, le précédent gouvernement a mis en place des mesures incitatives, comme le dispositif « Louer abordable ». Avec cet cet amendement, nous proposons d'aller plus loin, en exonérant de l'impôt sur la fortune immobilière- l'IFI -les personnes physiques dont les biens immobiliers sont mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants : conventionnement avec l'ANAH ou intermédiation locative. L'objectif est d'inciter les personnes physiques concernées par l'IFI à mettre en location leurs biens immobiliers dans le cadre des dispositifs solidaires et, ainsi, de favoriser le domaine locatif social.

Les dispositions proposées visent à compléter la composition de la CDAC, d'une part, par un représentant des maires des communes limitrophes au projet d'implantation et, d'autre part, par des représentants du tissu commercial, personnalités qualifiées en matière de commerce, d'artisanat,

elles présenteraient la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'effet du projet sur le tissu économique. Afin d'améliorer la prise en compte des impacts commerciaux des décisions des CDAC, il est proposé d'introduire, pour tout tout projet nouveau d'implantation commerciale, une obligation systématique d'audition par la CDAC des associations de commerçants et du manager de centre-ville de la commune d'implantation, lorsqu'ils existent. Enfin, il est proposé que les CDAC informent

qu'une recomposition de la CDAC serait l'alpha et l'oméga de la revitalisation des centres-villes me paraît complètement déconnecté de la réalité- je le dis tel que je le pense ! C'est un sujet qui nous oppose fortement et sur lequel

Il suffit de voir ce qui s'est fait depuis de nombreuses années pour être convaincu du contraire ! Pour moi, ce n'est absolument pas le coeur du sujet et, autant je crois avoir fait le

j'ai souhaité, dans le cadre de la revitalisation des centres-villes, que l'on puisse dans certains cas se passer de l'autorisation de la commission, ce n'est pas pour rien ! Je ne mets pas en doute l'honnêteté des personnes qui siègent

Là aussi, je dirai que le fonctionnement des CCI varie selon les personnes qui les président.

cosignée. Le présent article vise à modifier la composition des commissions départementales d'aménagement commercial, pour mieux représenter le tissu économique et les élus locaux. À cette fin, il intègre le maire d'une des communes limitrophes dans la composition de la CDAC, ce qui ne nous pose aucun problème. En revanche, il réintroduit au sein de la CDAC des acteurs économiques, au nombre de trois, désignés par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture, sans toutefois leur conférer le droit de vote. Afin de conserver le même nombre de membres et la répartition entre élus locaux et autres représentants, le nombre de personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, ainsi qu'en matière de développement durable et d'aménagement du territoire Cette modification, juridiquement contestable, est en infraction avec les règles européennes, comme nous l'a rappelé le rapporteur lors de la discussion de la proposition de loi Revitalisation. Ce dernier estimait ainsi qu'il était juridiquement délicat de faire de ces représentants consulaires des membres de cette commission, tant les intérêts sont mélangés, et ce quand bien même ces représentants siègeraient sans droit de vote. Nous estimons également que la juste représentation des consommateurs et des personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire

faire cesser ces activités commerciales sans autorisation, et les exemples se multiplient

Quel est l'avis de la commission ?

aux excellents experts que l'on trouvera sur tous les territoires, la CDAC disposera d'une vision à la fois complète et objective, qui lui permettra de rendre les meilleurs avis possible

qu'aucune friche existante ne permet l'accueil du projet qu'il envisage, en centre-ville, d'abord, puis en périphérie. Outre que la notion de friche n'est ni définie ni circonscrite, le choix d'une implantation répond à d'autres considérations, essentiellement commerciales.

La charge de la requalification des friches industrielles, administratives ou commerciales ne doit effectivement pas être supportée par le porteur d'un futur projet. En tout état de cause, l'établissement d'un nouveau commerçant est guidé par l'existence de flux de clientèle, et non par la seule disponibilité foncière,

encore qu'on nous ait tout à l'heure expliqué ce qu'il convenait de faire, parfois, de l'unanimité ... L'article 54 G, introduit en commission, instaure l'unanimité pour les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial remettant en cause un avis défavorable émis en commission départementale.

est déjà permise par l'article R.752-36 du code de commerce, ce qui rend inutile cet ajout.

prennent leur décision en fonction des dossiers qui leur sont soumis ? Ce n'est pas toujours le cas, et l'avis peut être fonction de ce qui se passe sur le terrain. La situation, comme je l'ai dit, est diverse selon les territoires.

la DGCCRF estime ne plus disposer de moyens humains pour agir. Dans le même temps, cela a été dit, des milliers de mètres carrés sont construits tout à fait illégalement, au grand dam des élus.

pour examiner directement, sans examen préalable par les commissions départementales, les demandes d'autorisation en vue d'ouvrir des surfaces de vente supérieures à 20 000 mètres carrés. Cela représente à peu près une dizaine de dossiers par an. depuis 2015, la Commission nationale utilise systématiquement son pouvoir d'autosaisine, soit pour émettre un avis, soit pour rendre une décision sur la conformité de ces projets par rapport aux critères de l'article L. 752-6 du code de commerce. présente deux avantages notables. D'abord, elle permettra de gagner du temps, environ cinq mois. Ensuite, l'instruction de la demande offrira les mêmes garanties, s'agissant de l'impact local du projet, puisque la composition de la Commission nationale sera complétée par les élus locaux membres de la commission départementale. Enfin, pour les projets importants, le délai d'instruction reste bref, puisque, au-delà de quatre mois à compter de la saisine, l'avis ou la décision de la Commission nationale sont réputés favorables. Par ailleurs, cet amendement répond à l'attente des professionnels des centres commerciaux des centres-villes et de la périphérie, des centres à thèmes ou des nouveaux parcs d'activités commerciales. Ne l'oublions pas, ce sont des acteurs majeurs de la vie économique et sociale de nos territoires, car ils représentent près de 450 000 emplois non délocalisables et génèrent, sur un chiffre d'affaires annuel de 118 milliards d'euros, 25,5 milliards d'euros de taxes et d'impôts par an. Quel

vigueur imposait une autorisation d'exploitation commerciale pour créer un magasin par transfert d'une activité existante ou pour réutiliser à usage de commerce de détail un local appelé à être libéré. La loi précitée a supprimé la notion de transfert, ce qui a entraîné deux conséquences. D'abord, le commerçant doit déposer un projet de création soumis à autorisation. Ensuite, le local libéré peut être commercialisé de nouveau sans être soumis à une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, sauf dans deux cas

Il nous faut donc réintroduire dans la loi la notion d'autorisation de création par transfert, afin d'assurer la réhabilitation des entrées de ville, à charge pour le pouvoir réglementaire de préciser clairement la liste des pièces complémentaires à joindre au dossier de demande pour que le pétitionnaire justifie

cette notion dans la loi qui pourrait doublonner avec d'autres cas d'ouverture. Quant à la question de l'harmonisation des approches des CDAC en la matière, elle est réelle, mais il n'est pas évident que la modification proposée soit de nature à la résoudre.

entrer en contradiction avec une autre disposition de l'article L. 752-1 du code de commerce qui permet la reprise, sans autorisation de la commission, d'un local d'une surface de vente de plus de 1 000 mètres carrés délaissé depuis moins de trois ans après exploitation, sous bénéfice d'une autorisation.

Enfin, il soumet à autorisation les entrepôts de e-commerce d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. Ces mesures restrictives, qui élargissent le champ des autorisations obligatoires de la commission, modifient les équilibres que nous essayons de trouver entre liberté du commerce et redynamisation des centres-villes, y compris hors ORT. les seuils des projets soumis à autorisation à l'échelle nationale entraînera des conséquences importantes, y compris sur l'organisation et l'efficacité des CDAC, qui ne sont, en tout état de cause, pas outillées pour répondre à une telle augmentation des dossiers. Une augmentation

d'un permis de construire, hormis à Paris, qui a expérimenté un seuil à 400 mètres carrés, pourrait être très important dans certains territoires. Les CDAC ne sauraient y faire face sans dégrader l'instruction de l'ensemble des dossiers. J'ajoute que, dans le cadre de la législation actuelle, les communes de moins de 20 000 habitants peuvent déjà solliciter la CDAC pour l'examen des projets de moins de 1 000 mètres carrés.

effets de la suppression de l'autorisation en centre-ville qui est l'un des éléments forts du projet que nous portons dans l'intérêt de la redynamisation des centres-villes.

de rétablir un passage en CDAC. Telles sont les raisons pour lesquelles je demande à la Haute Assemblée d'adopter cet amendement de suppression. Quel est l'avis de la commission ? Cette disposition

à 500 mètres carrés à l'égard des ensembles commerciaux mentionnés à l'article L. 752-3 du code de commerce. Ces ensembles commerciaux peuvent en effet être constitués de plusieurs commerçants indépendants qui n'exploitent qu'un espace de vente d'une superficie réduite, souvent très inférieure au seuil de 500 mètres carrés. Certains sont du reste parfois les producteurs eux-mêmes ils trouvent dans ce type de surface commerciale un lieu de vente pour leur propre production. Le maintien à 1 000 mètres carrés du seuil d'intervention de la CDAC

Il offre aux maires, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, la possibilité de déroger à certaines normes environnementales ou d'accessibilité. Ainsi, le maire d'une commune signataire d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire pourra demander au représentant de l'État dans le département de déroger aux normes précitées. mes chers collègues, l'acceptation d'une telle disposition contribuera à une application disparate sur le territoire national des règles environnementales et d'accessibilité.

Le Gouvernement a bien sûr injecté 5 milliards d'euros dans la corbeille pour revitaliser 222 villes sur les 700 qui se trouvent en difficulté. Si nous voulons simplement doubler la mise pour que quelque 220 villes supplémentaires soient prises en compte, il faudrait 1 milliard d'euros supplémentaire par an. C'est ce que nous avions

du commerce adaptées aux spécificités de chaque territoire. En attribuant aux communautés de communes et d'agglomération une compétence « politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt communautaire », la loi NOTRe a ouvert un renouveau de la gouvernance locale de cette problématique à l'échelle intercommunale et à l'élaboration de stratégies commerciales territoriales. Cet amendement vise à encourager et à accélérer ces évolutions en responsabilisant davantage les territoires : il s'agit de permettre aux intercommunalités de décider des règles applicables en matière d'implantation commerciale, dès lors qu'elles peuvent attester de l'élaboration d'une stratégie commerciale, de la mise en place d'une gouvernance locale adaptée, d'une politique active d'animation du tissu économique local et de l'instauration d'un système local d'observation pérenne des dynamiques commerciales.

Nos acteurs locaux, libérés de cette taxe, pourraient être incités à choisir des matériaux plus esthétiques et innovants pour embellir leur devanture. À travers ce mécanisme d'incitation, nous restons donc cohérents avec les objectifs fixés par la Haute Assemblée, à savoir la revitalisation

Simplifier et libérer les petits commerces d'une contrainte fiscale supplémentaire tout en embellissant notre cadre de vie, telle est la volonté que nous exprimons à

Pourtant, celle-ci est étroitement liée au logement et aux situations de précarité en général. Selon l'Observatoire national de la précarité énergétique, l'ONPE, elle touche près de 5 millions de ménages en France, soit 12 millions d'individus.

Or pouvoir se chauffer, s'éclairer, cuisiner, chauffer l'eau pour se laver ne doit pas devenir un luxe. L'énergie est un droit pour toutes et tous, et c'est une nécessité de la vie quotidienne. Pour cette raison, nous sommes contre les coupures, qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité ou du gaz, y compris hors de la trêve hivernale. Nous sommes pour un service public de l'énergie

se déroulent chez Engie, Enedis, et GRDF ; je pense aux plans sociaux en cours et aux délocalisations d'emplois déjà externalisés ; je pense au silence des directions et au relatif silence des médias- il ne faudrait surtout pas souffler sur les braises de la contestation Ce mouvement social traduit un élan : celui de salariés qui demandent ce service public de l'énergie, qui passent des usagers en heures creuses ou rouvrent des agences EDF, comme à La Courneuve ou à Ivry.

puissent se référer à une année de consommation énergétique permettant la prise en compte de références fiables ou disponibles. Or les données de 2010 ne le sont probablement plus. Ainsi, il serait possible d'inclure un bâtiment, public ou privé, construit après 2010 et n'ayant pas fait l'objet d'un référentiel de consommation. Quel est l'avis de la commission ?

lorsque des actions de réduction de la consommation d'énergie ont été menées avant cette date. Ainsi, il serait possible d'inclure les propriétaires de bâtiments ayant engagé des travaux en vue de baisser la consommation énergétique, notamment les créés par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de juillet 2005. Les objectifs resteraient inchangés pour chacune des échéances fixées, en 2030, 2040 et 2050.

. Le présent amendement vise à faire figurer les surfaces parmi les critères de modulation, en plus du changement d'activité ou du volume d'activité. Selon l'exposé des motifs du présent projet de loi, « il est proposé d'acter le principe d'un objectif de modulation voire de dispense selon la taille du bâtiment, un immeuble de bureau disposant de plus de moyens qu'un petit commerce de proximité. » Il importe que les critères de modulation incluent également les surfaces des bâtiments concernés. En effet, si la surface figure dans les déterminants du décret, elle n'est pas citée parmi les éléments énumérés au I de

mais aussi le potentiel de réduction propre à chaque activité. Il convient également de prendre en compte les changements d'usage qui ne correspondent pas à un changement d'activité.

de loi prévoit déjà que les objectifs peuvent être modulés en fonction de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale. Il convient néanmoins de prendre en compte les montants en jeu, et non la santé financière de l'entreprise ou de la collectivité territoriale concernée. Cet amendement vise à faciliter la mise en oeuvre des actions de réduction des consommations énergétiques, dans l'hypothèse où la situation financière de l'assujetti ne lui permettrait pas d'assumer les charges liées aux travaux nécessaires. Quel est l'avis de la commission ? L'adoption

de sa situation financière ? Je rappelle que le projet de loi permet de moduler l'obligation en cas de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus. En outre, la commission a supprimé toute sanction

en fonction de la part d'énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d'énergie finale. Le développement des énergies renouvelables contribue en effet à réduire la dépendance énergétique de la France et les émissions de gaz à effet de serre.

d'introduire un critère de modulation des objectifs relatifs à la part des énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d'énergie finale.

les réseaux collectifs en énergies renouvelables. Nous proposons de corriger les effets collatéraux d'objectifs exprimés désormais en énergie finale et non plus en énergie primaire.

en quelques mots sur l'importance des réseaux de chaleur. Un réseau de chaleur dans une collectivité, quelle qu'elle soit, permet, en jouant sur des économies d'échelle, d'obtenir des effets importants en termes de réduction de la consommation d'énergie et de verdissement des énergies. Je pense donc qu'il y a erreur d'analyse. Peu importe, le combat continue : je continuerai de le mener, parce que c'est un enjeu important pour notre pays

: La parole est à M. Guillaume Gontard. L'article 55 traite des enjeux de rénovation énergétique pour les bâtiments tertiaires et précise les modalités d'application de cette obligation. L'article 17 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte précise cette obligation en la prolongeant par périodes de dix ans entre 2020 et 2050, avec un niveau de performance fixé pour chaque décennie, afin d'aboutir à une réduction des consommations d'énergie finale du parc concerné d'au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010.

Il est ainsi prévu d'obliger les propriétaires ou les locataires de certains bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire à mettre en oeuvre des actions de réduction de la consommation d'énergie pour arriver à une diminution des consommations d'énergie de l'ensemble de ces bâtiments d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010,

En effet, au-delà de la volonté de réduire la consommation d'énergie finale, il convient de mener une politique incitative sur le matériel de production, en encourageant la transition de celui-ci vers des énergies renouvelables à faibles émissions de CO2. Nous proposons donc que, en cas de changement de matériel de production énergétique, l'alternative en énergies renouvelables soit étudiée par le propriétaire par comparaison avec une solution en énergies carbonées. Cet amendement sert l'objectif ambitieux et nécessaire de l'article que nous examinons. Quel est l'avis de la commission ? Il ne me l'avis de la commission ? Il ne me semble pas opportun d'ajouter une telle obligation. Il est préférable que les assujettis consacrent leurs sommes disponibles à engager des actions pour réduire leur consommation plutôt qu'à réaliser des études pour changer leurs sources d'alimentation.

Notre collègue Gontard a rappelé les données de la trajectoire d'économies d'énergie à réaliser d'ici à 2050

que les propriétaires d'un patrimoine important, c'est-à-dire de plusieurs bâtiments, aient l'obligation de lancer, d'ici à 2030, une réflexion sur les possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique. Instaurer

Les modalités de cette évaluation seraient précisées dans le décret déjà prévu au III de l'article 55. Ces études pourraient être financées par des certificats par des certificats d'économies d'énergie. Elles paraissent saines si l'on veut tenir cette trajectoire, et nécessaires pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans les étapes successives qui ont été prévues.

à celui de la commission. Le projet de loi fixe un objectif de résultat, en visant à la responsabilisation des acteurs et en excluant la prescription d'objectifs de moyens. C'est d'ailleurs ce que nous soutenons de manière générale, s'agissant en particulier des questions normatives- j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises quel est sur ce point l'objectif du Gouvernement. Il nous paraît beaucoup plus opérationnel de laisser le choix aux acteurs et de ne pas imposer par la loi un audit qui s'avère souvent coûteux. Certains acteurs opteront pour des audits globaux, d'autres réaliseront des travaux d'amélioration, de maintenance ou des actions de sensibilisation des occupants. de ces amendements forcerait à réaliser un nouvel audit certains assujettis qui en auront déjà produit un avant l'entrée en vigueur de la loi. De plus, certains bâtiments du secteur tertiaire sont d'ores et déjà soumis à l'obligation

Une grande majorité des propriétaires de ces parcs dans le domaine tertiaire sont soucieux d'entretenir leur patrimoine. En revanche, nous constatons qu'il y a de véritables passoires énergétiques, parce qu'une partie des propriétaires cherchent

l'amendement n° 124 rectifié . Nous proposons de préciser que l'usage des bâtiments sera pris en compte dans la détermination par décret des catégories de bâtiments soumis à l'obligation, en complément de la surface et du type d'activité exercée à titre principal.

agréées. De même, il convient d'instaurer une procédure de sanction en cas de non-respect des obligations prévues par l'article 55, afin que les bâtiments tertiaires atteignent réellement les objectifs de réduction des des consommations d'énergie. Tel qu'il est rédigé aujourd'hui, le décret ne prévoit pas une telle procédure. Quel

peu compréhensible, une sanction administrative qui ne concernerait que ceux qui choisiraient la première branche de l'alternative. Ensuite, en matière de rénovation des bâtiments, la commission juge préférable de mener des politiques incitatives,

sans sanction administrative au contrôle avec sanction administrative. Le secteur de l'immobilier tertiaire se caractérise par une sanction du marché qui affecte la valeur du bien. Par ailleurs, deux modalités sont déjà prévues dans le dispositif : une obligation de transmission d'informations qui caractérisent le respect des économies d'énergie, en annexe à la promesse ou au compromis de vente ou, en cas de location, au contrat de bail, et la publication par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent des consommations énergétiques au cours des trois dernières années écoulées, des objectifs passés et de l'objectif à venir. Nous ne souhaitons pas instaurer à ce stade une autre forme de sanction, qui pourrait être perçue comme une obligation nouvelle.